La séance est reprise. Nous poursuivons la discussion du projet de loi relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique.

Les articles 64 et 66 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite « loi NOTRe », ont rationalisé l'exercice des compétences en matière de gestion touristique, en introduisant dans le code général des collectivités territoriales la « promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme » parmi les compétences obligatoires des communautés de communes et des communautés d'agglomération, transférées au plus tard le 1 janvier 2017. de coopération intercommunale, les EPCI, ont aujourd'hui la priorité pour l'institution de la taxe de séjour, et que la condition de leur éligibilité est « la réalisation d'actions de promotion en faveur du tourisme ». Ces actions étant de la compétence de leur office de tourisme, la taxe de séjour est par conséquent collectée par l'EPCI. Cette dernière est destinée « à favoriser la fréquentation touristique du territoire Elle est généralement affectée au financement des actions de l'office de tourisme, de manière obligatoire si ce dernier est un établissement public industriel et commercial, Je rappelle que déjà, à l'époque, l'application de la loi NOTRe avait suscité une vive inquiétude parmi les maires de communes touristiques, inquiétude relayée par ailleurs dans ce même hémicycle. Aujourd'hui, en Martinique, les maires dénoncent ces dispositions qui appauvrissent, financièrement et touristiquement, leur commune. Ils dénoncent la régression des politiques touristiques dans la majorité des communes de Martinique. Je rappelle qu'aucune commune de Martinique ne dispose du label « station de tourisme » eu égard aux conditions requises pour l'obtenir. C'est pourquoi ils ont demandé aux parlementaires que nous sommes d'intervenir afin de leur permettre de récupérer cette prérogative, dans l'intérêt de leurs communes. Je considère également, monsieur le ministre, qu'il est urgent d'organiser une réunion de travail avec les municipalités locales, pour remédier à ce problème d'importance. Mme Michelle Gréaume. Par cet amendement, nous proposons de rendre la compétence « promotion du tourisme, dont la création d'offices du tourisme » facultative, alors qu'actuellement elle est obligatoirement transférée aux EPCI, afin que toutes les communes puissent bénéficier de nouveau de cette compétence et décider librement de son transfert ou non. Encore une fois, nous estimons que le texte ne va pas assez loin et rompt l'égalité entre les communes. La promotion du tourisme, et notamment la gestion de l'office du tourisme, est importante pour les communes et fortement liée à leur image. Le transfert rendu obligatoire par la loi NOTRe de cette compétence vers les EPCI a eu un lourd impact sur les communes. Permettre aux seules communes classées « stations de tourisme » de récupérer cette compétence pénalise de nombreuses communes, auxquelles ce classement aux critères méticuleux a été refusé ou qui n'ont pas pu assumer les tâches administratives relatives à la présentation d'un tel dossier.

M. Jean-Marc Gabouty. Cet amendement a pour objet d'étendre à toutes les communes touristiques la possibilité de retrouver l'exercice de la compétence « tourisme ». L'article 6 restreint cette possibilité aux seules communes touristiques reconnues stations classées de tourisme, ce qui crée une différence de traitement de traitement injustifiée entre communes touristiques. Toutes ces communes devraient en effet pouvoir choisir librement l'organisation touristique la plus adaptée à leur situation : exercer leur compétence et conserver un office de tourisme communal, ou la transférer de façon volontaire au niveau intercommunal. Le modèle intercommunal peut se révéler inadapté à certaines communes touristiques, par exemple lorsqu'elles sont dissoutes dans un ensemble de collectivités n'ayant pas les mêmes orientations touristiques. Elles n'ont alors aucune marge de manoeuvre pour défendre leurs intérêts touristiques propres et sont donc privées du pouvoir de mener à bien une stratégie appropriée. Les spécificités des 1 900 communes touristiques peuvent nécessiter de conserver un pilotage de leur promotion et une gouvernance au plus près des réalités locales. Cet amendement vise à leur permettre de retrouver les marges de manoeuvre nécessaires. L'amendement

Cet amendement vise à donner davantage de liberté aux acteurs locaux pour définir les modalités d'organisation de la compétence promotion du tourisme. En effet, l'exercice concomitant de la même compétence par deux acteurs sur le territoire de la commune peut être source de difficultés. Aussi, l'amendement a pour objet qu'un accord soit conclu entre la commune et l'EPCI, afin que, au cas par cas, les afin que, au cas par cas, les acteurs locaux s'accordent sur la manière la plus pertinente de déployer cette politique.

Cette décision fragilisera des ensembles qui ont été mis en place et commencent à fonctionner. C'est tout ce que

est une autorité nommée en conseil des ministres : il est donc une autorité nationale déconcentrée. Tant pis si certains pays dans le monde ne comprennent pas ce qu'est l'institution préfectorale. Pour ma part, je considère que Franck Robine, préfet de la région Martinique, sera toujours mieux placé

le souci de nos communes classées de ne pas laisser galvauder un label national qu'elles ont conquis de haute lutte,

émis un avis défavorable, que je réitère. La parole est à M. le ministre. Puisque nous sommes à une heure avancée, monsieur le président de la commission des lois, permettez-moi de vous confier un secret. Le ministre chargé du tourisme suit l'autorité préfectorale. En tout cas, il ne viendrait pas à l'esprit d'un ministre normalement constitué de passer outre pour de mauvaises raisons- vous avez d'ailleurs Je vous propose collectivement, puisque nous sommes des militants de la proximité, d'y faire droit de manière très concrète dans ce cas de figure. Au fond, s'agissant de la signature préfectorale,

d'un pouvoir central, puisque c'est de la déconcentration. On n'abîme pas ce label, il n'est pas galvaudé, précisément parce que les autorités préfectorales y veillent. En tout cas,

que les soi-disant passe-droits accordés ne le seront qu'avec une grande modération, en ne réglant que des situations extrêmement prégnantes qui peuvent développer le tourisme dans nos territoires, particulièrement en outre-mer.

il est vrai que nous obéissons à un régime un peu particulier -, ont été transférées aux territoires. Je voudrais aussi rappeler que l'Île-de-France est une région

pour objectif de redonner, bien sûr, de la souplesse et de la liberté, et surtout de permettre aux maires de choisir les compétences qu'ils souhaitent ou non exercer.

et la proximité. C'est totalement incompréhensible. Aujourd'hui, monsieur le ministre, vous le savez, le pays ne va pas très bien, il est dans une situation assez préoccupante. Votre intérêt, vous l'avez compris, c'est de vous appuyer sur les communes

un grand mérite, ainsi que les amendements qui suivent : il tend à partir d'un diagnostic que je crois juste. En effet, dans un certain nombre de cas, il est souhaitable que, compte tenu de la taille d'une intercommunalité, il puisse

les Hauts-de-Seine. En effet, il faut un nombre suffisamment important de communes qui demandent à avoir leur propre plan au sein de l'intercommunalité pour que cette faculté puisse être mise en vigueur. Évidemment, dans les Hauts-de-Seine, il n'y aura jamais suffisamment de communes pour faire plusieurs plans locaux d'urbanisme à l'intérieur d'une intercommunalité de la métropole du Grand Paris.

pour le cas particulier qui est le vôtre, cette disposition rétroagirait sur l'ensemble des départements qui sont dans une situation différente, au risque même de rendre très difficile l'élaboration de plans locaux d'urbanisme intercommunaux là où ils seraient nécessaires. C'est pourquoi je voudrais en toute sincérité vous inviter à retirer votre amendement pour que nous puissions le retravailler, afin d'examiner à quelles conditions il pourrait être fait droit à votre préoccupation, sans pour autant qu'il y ait ces effets induits sur des départements qui, disons-le, auraient un caractère plus rural que le vôtre. Comme je sais que vous êtes vous-même de cette France des territoires ruraux, vous comprendrez le point de vue que j'ai essayé de vous exposer. C'est la raison pour laquelle la commission des lois, après en avoir là aussi longuement délibéré, vous serait très reconnaissante de bien vouloir retirer votre amendement. Quel est

tout est fait non seulement pour achever la carte intercommunale, quitte à tordre la volonté des petites communes en particulier en milieu rural, mais également pour renforcer les transferts de compétences à l'échelon intercommunal en matière d'aménagement du territoire. C'est ainsi que la loi portant engagement national pour l'environnement a permis la reconnaissance et favorisé l'essor des PLU intercommunaux. La loi ALUR, en allant plus loin, a rendu ce transfert obligatoire, sauf minorité de blocage. Cette évolution a entraîné de nombreuses difficultés sur le terrain, puisque nombre d'élus se sont trouvés coincés dans des intercommunalités qu'ils n'avaient pas choisies, où le transfert de compétence s'est opéré sans leur accord et dont l'adoption a été également permise sans leur accord. Que reste-t-il alors à ces élus comme outil de maîtrise de leur territoire ? C'est une véritable question Pour cette raison, notamment, ce projet de loi a allégé et « adouci » ces transferts de compétences obligatoires pour remettre de la souplesse dans la construction intercommunale. Nous en prenons acte et partageons cette volonté. Pour autant, et parce qu'il Pour autant, et parce qu'il s'agit d'une problématique très spécifique, celle de la réalisation d'un plan local d'urbanisme, qui délimite à la parcelle l'affectation des sols, nous considérons qu'il convient d'être plus ambitieux dans le respect de la volonté communale. Soyons clairs, lorsque les communes le désirent, par un transfert de compétence librement consenti, il est intéressant de disposer de ce type de document au niveau intercommunal- personne ne le conteste. Pour autant, ce qui est souhaitable ne doit pas devenir forcément obligatoire. Nous proposerons donc des amendements qui, à chaque étape de la réalisation de ce document, du transfert de compétence à son adoption, tendent à faire respecter la volonté des communes membres de l'intercommunalité.

Mais en réalité si toute compétence en matière d'aménagement et de réalisation d'un plan local d'urbanisme, outil premier d'un projet municipal, est ôtée à ces élus et ces équipes nouvellement élues, c'est une nouvelle fois

ont été définies dans la loi ALUR en 2014 pour les communautés de communes et d'agglomération. Deux options leur étaient alors proposées : soit le transfert de la compétence pouvant se faire de manière volontaire jusqu'au 27 mars 2017, soit le transfert soit le transfert de plein droit, sauf si une petite minorité s'y opposait- 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population totale des communes concernées. En réalité, en cas d'objection, seul un report de transfert au 1 janvier 2021 était prévu. La collectivité n'a donc pas eu son mot à dire. C'est sur ce point qu'il s'agit de redonner un droit de parole aux maires, et pas simplement lorsque le PLUI est déjà inscrit sur leur territoire, comme le prévoit l'article 7. Cet amendement vise à conditionner l'élaboration intercommunale d'un PLU à un transfert volontaire et explicite à l'EPCI de la compétence « PLU » par la commune. Chaque maire, dans chaque commune, devrait pouvoir choisir de déléguer l'établissement de l'ensemble des normes applicables à l'utilisation du sol de son territoire à l'intercommunalité. Ce n'est qu'à cette condition que les communes et leurs maires pourront être véritablement associés à l'élaboration d'un PLU. Quel est l'avis de la commission Merci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

d'agglomération. L'effet de ces amendements serait contraire à l'objectif, puisque la compétence liée au PLU demeurerait inscrite dans les compétences obligatoires de ces catégories d'EPCI. Serait cependant supprimée la possibilité pour une minorité de communes de s'opposer au transfert de ces compétences.

PLUI. Toutefois, ce dispositif pourrait concrètement se réduire à une simple consultation formelle, sans prise en compte réelle de l'avis formulé. Cet amendement a pour objet d'aller un cran au-dessus pour tenir compte de l'avis des communes membres de l'EPCI : il s'agit d'obliger le président de celui-ci à informer les communes des raisons précises qui ont conduit à ne pas respecter l'avis des communes. Cette justification précise nous semble accroître

car, dans les faits, le principe de consultation revêt trop souvent la forme d'une simple formalité administrative, au lieu de donner lieu à des échanges constructifs avec l'EPCI. Les maires sont ceux qui connaissent le mieux leur commune, et il est tout à fait logique qu'ils puissent se faire entendre par leur EPCI. En amenant celui-ci à expliquer les raisons précises de sa décision, cette proposition va dans le sens de la concertation entre les acteurs publics. Elle favorise donc une meilleure coopération intercommunale basée sur l'échange et le dialogue., ce dispositif aurait pour conséquence une meilleure transparence de l'action publique

pour tenir compte de l'avis de la commune. À défaut, c'est-à-dire en cas d'avis défavorable de la commune sur la modification en question, la majorité des deux tiers reste nécessaire. Cet article, si nous en jugeons positive l'intention, ne change en réalité pas grand-chose, puisqu'en cas de désaccord de la commune, la règle des deux tiers est maintenue. Nous estimons pour notre part, et alors que le PLU est un document programmatique majeur de la vie démocratique locale, traçant le projet de ville pour de nombreuses années, que l'accord des collectivités composant l'intercommunalité à la manoeuvre n'est pas négociable. n'est pas négociable. Ainsi, dans un contexte où nombre d'intercommunalités sont non pas choisies, mais subies, qu'en milieu rural elles regroupent un nombre très important de communes, le respect de l'échelon local doit être la règle. Pour traduire cette exigence, nous proposons que le projet de PLU ne puisse être adopté tant qu'une commune émet un avis défavorable sur le règlement ou les orientations relatives au territoire la concernant. Le respect de la démocratie locale et de la légitimité démocratique est à ce prix.

ne doit pas rester qu'une simple formalité. Cet avis doit être réellement pris en compte et les raisons précises qui ont conduit à ne pas respecter l'avis des communes dans le PLUI doivent être clairement transmises à ces dernières ? Comme pour l'amendement n° 762, si leur position n'est pas prise en compte, elles doivent en revanche savoir précisément pour Cela contribue à créer un climat de confiance dans un contexte où, dans de nombreuses municipalités, le transfert à l'EPCI de la compétence « PLU » a été plus ou moins mal vécu.

la prise en compte, comme cela a été dit, de l'avis des communes sur les plans de secteur qui couvrent leur territoire, en obligeant l'EPCI à justifier la non-prise en compte de l'avis. Cette nouvelle procédure serait redondante avec la demande d'avis de l'ensemble des communes sur le projet de PLUI, à la suite de laquelle le plan

les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d'enquête aient été présentés lors d'une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l'EPCI. Il s'agit d'un dossier majeur pour le territoire, je vous propose de prévoir la présence des maires délégués au sein de la conférence intercommunale au cours de laquelle seront présentés les avis, les observations et le rapport. ? Cet amendement vise à associer les maires délégués à la conférence intercommunale qui se réunit au début et au terme de la procédure d'adoption d'un PLUI.

Merci Dans le cadre des procédures de modification ou de modification simplifiée des plans locaux d'urbanisme, aucun délai n'encadre la réception des avis des personnes publiques associées, les PPA, après que le dossier leur ait été notifié. Pourtant, lors de la phase initiale d'élaboration du plan local d'urbanisme, les PPA disposent d'un délai de deux mois pour rendre leur avis. En effet, à défaut de réponse des personnes publiques associées dans les huit semaines suivant l'envoi du projet, elles sont réputées favorables au PLU. Dans le cadre d'une modification ou d'une modification simplifiée, faute de délai, les avis des PPA peuvent arriver tardivement lors de l'enquête publique. Or ces avis doivent être joints au dossier d'enquête publique. Ce défaut d'encadrement des délais de réponse des personnes publiques associées est un moyen régulièrement soulevé lors des recours sur les procédures de PLU,

des seuls avis émis. La procédure simplifiée prévoit, elle, que les avis qui sont, le cas échéant, remis par les personnes publiques associées sont mis à la disposition du public.

M. le président de la commission de mon soutien plein et entier aux assouplissements proposés aux communes membres des établissements publics de coopération intercommunale. Je considère que ces propositions permettront de donner plus de latitude aux communes et plus de voix à leur maire. En revanche, comme nous pouvons l'observer depuis mardi au fil des différents débats, donner plus de liberté ne doit pas se traduire par une généralisation à toutes les échelles d'outils qui sont voués à répondre à des problématiques locales de proximité. Ainsi, il nous paraît cohérent de ne pas toucher aux dispositions actuellement en vigueur pour les métropoles et pour les communautés urbaines. C'est le sens de cet amendement, qui vise à créer une exception excluant ces dernières du dispositif. En France, métropoles et communautés urbaines sont le plus souvent de grandes villes, anciennement Pour ces EPCI, l'urbanisme doit nécessairement se concevoir à plus grande échelle. Dans leur cas, la continuité urbaine ne s'arrête pas aux limites entre chaque municipalité. Par la force des choses, la pratique du document d'urbanisme à l'échelle intercommunale a une histoire plus longue

La procédure de modification simplifiée des PLU impose deux délibérations : la première doit définir les modalités de mise à disposition du public ; la seconde, en fin de procédure, doit approuver le document modifié. Il est possible d'éviter la première délibération en définissant les modalités de mise à disposition du public par arrêté du président. Notons que la procédure de modification de droit commun comporte une seule délibération. En effet, les modalités de l'enquête publique sont justement définies par un simple arrêté du président.

L'article 7 du projet de loi permet à un maire de prendre

notre collègue François Bonhomme propose, dans le cas d'une modification simplifiée, que ce soit le président de l'EPCI ou le maire, et non l'organe délibérant de l'EPCI ou le conseil municipal, qui définisse les modalités de mise à disposition du public. La procédure de modification simplifiée étant rapide, la double délibération de l'EPCI

intercommunale imposent souvent un plan local d'urbanisme intercommunal aux communes et la loi a lié le transfert du plan local d'urbanisme vers les EPCI à celui du droit de préemption urbain, Cet amendement a pour objet de dissocier le PLUI du DPU exercé par les établissements publics de coopération intercommunale. Dans certains EPCI, le PLU a été transféré des communes vers l'intercommunalité, privant de manière stricte et trop rigoureuse les communes du DPU. L'argument avancé en faveur du transfert de la compétence- automatique dans le cas des métropoles et des communautés urbaines, facultatif dans le cas des communautés d'agglomération et des communautés de communes -est fallacieux, car il confond la planification d'urbanisme, dont l'EPCI peut être la bonne échelle, et l'urbanisme opérationnel, qui peut être conservé par les communes membres. Il en résulte une frustration légitime de beaucoup de maires, qui souhaiteraient conserver les outils de l'urbanisme opérationnel. l'amendement vise à renforcer le principe de subsidiarité, en redonnant à la commune la compétence du DPU de plein droit, tout en conservant la faculté, pour le conseil municipal, de déléguer cette compétence à l'EPCI. Les différentes communes d'un même EPCI pourraient ainsi conserver le DPU sans pour autant remettre en cause les stratégies intercommunales de planification d'urbanisme.

de dissocier l'aspect de planification, lié au PLUI, et l'aspect d'urbanisme opérationnel, attaché à l'exercice du droit de préemption. L'exercice du droit de préemption nécessite une connaissance fine du territoire et ne peut se faire que dans l'ultra-proximité. La commission émet donc un avis favorable

de la compétence PLU pour l'ensemble des établissements de coopération intercommunale. Le Sénat avait alors imposé, dans la discussion avec le Gouvernement, l'instauration d'une minorité de blocage, fixée à 25 % des communes, représentant au moins 20 % de la population. Nous avions, à l'époque, soutenu ce qui nous semblait un compromis acceptable, en considérant que la suppression pure et simple de la disposition, que nous proposions, ne passerait pas le stade de l'examen par l'Assemblée nationale. La position du Sénat avait alors prévalu et été maintenue jusqu'en commission mixte paritaire. Pour autant, alors que plusieurs années ont passé et que l'achèvement de la carte intercommunale s'est fait au forceps, à défaut et parfois même à revers de la volonté des communes, il convient de revenir sur ces transferts de compétences automatiques, l'existence d'une simple minorité de blocage n'étant pas suffisante. Ainsi, le PLU étant un document particulièrement sensible, les communes doivent pouvoir choisir de déléguer ou non la compétence liée à la réalisation de ce document d'urbanisme. Nous ne pouvons traiter le PLU comme un banal document : il s'agit de l'outil premier de mise en oeuvre d'un projet politique sur un territoire. Le projet d'aménagement et de développement durable définit les enjeux de développement et indique les objectifs afin d'y répondre,

enrôlées dans des intercommunalités « XXL » subies, car délimitées par le préfet, se voient privées contre leur gré de cet outil d'aménagement très fin et précis. Une telle situation nous semble particulièrement inacceptable, car elle reviendrait sur la capacité des élus municipaux à mettre en oeuvre le programme sur lequel ils ont été élus et qui a été soutenu par la majorité de la population. Nous proposons donc, par cet amendement, de revenir sur les transferts automatiques de compétences liés au PLU.

Cet amendement vise à reporter la date prévue de caducité des plans d'occupation des sols au 31 décembre 2019 dans les communes membres d'une intercommunalité qui n'aurait pas achevé son plan local d'urbanisme intercommunal. La loi ALUR a fixé au 31 décembre 2019 la caducité des POS d'une commune, à condition que l'EPCI ait prescrit l'élaboration d'un PLUI avant le 31 décembre 2015. Un certain nombre d'intercommunalités n'auront pas achevé leur plan local d'urbanisme avant le 31 décembre 2019, entraînant l'application du règlement national d'urbanisme, le RNU, ce que redoutent les communes concernées. Ainsi, 1 102 communes disposaient encore d'un POS opposable au 31 décembre 2018 dans le cadre d'une procédure d'élaboration de PLUI. C'est d'autant plus problématique pour ces communes pour ces communes qu'elles ne maîtrisent pas le calendrier d'élaboration du PLUI. Ainsi, elles risquent d'être pénalisées pour une situation dont elles ne sont pas responsables. Cet amendement vise à reporter au 31 décembre 2020

d'abord imaginé un autre mécanisme, mais, après réflexion avec les rapporteurs, je vous propose finalement de reprendre l'article 24 de la proposition de loi relative à l'équilibre territorial

voilà un bon amendement, que vous n'avez pas de raison de refuser ! Il s'agit de redonner aux communes la possibilité de garder la compétence des opérations d'aménagement et de mise en oeuvre des projets urbains. Je propose de rendre des pouvoirs d'urbanisme aux maires, qui sont aujourd'hui asphyxiés et paralysés par l'enchevêtrement des normes et qui ne peuvent plus rien faire. Merci, mes chers collègues, de soutenir ce bel amendement ! Quel est l'avis de la

la commune ne peut plus intervenir en matière de ZAE, en raison de la suppression de l'intérêt communautaire, ces zones relevant désormais uniquement des communautés.

devant faire l'objet d'un transfert obligatoire ; d'autre part, la divergence des services de l'État quant à l'approche globale et intégrée de cette compétence soulève des difficultés pour déterminer les contours de cette compétence. Ainsi, le rétablissement de l'intérêt communautaire redonnerait aux communes la liberté de décider des ZAE pour lesquelles l'échelon communautaire serait le plus pertinent et de celles qui pourraient rester dans le giron communal.

d'autre part, la divergence des services de l'État quant à l'approche globale et intégrée de cette compétence soulève des difficultés pour déterminer les contours de cette compétence. Ainsi, le rétablissement de l'intérêt communautaire pourrait redonner aux communes une liberté de décider des zones d'activités économiques pour lesquelles l'échelon communautaire serait le plus pertinent et de celles qui pourraient rester dans le giron communal. J'ajoute que j'avais déjà saisi déjà le ministre de l'intérieur en mars 2018 à ce sujet ; il m'avait

Merci,

D'une part, il n'existe pas de définition législative ou jurisprudentielle permettant d'identifier les zones d'activité économique devant faire l'objet d'un transfert obligatoire. D'autre part, la divergence des services de l'État quant à l'approche globale et intégrée de cette compétence soulève également des difficultés sur la détermination des contours de cette compétence. Ainsi, le rétablissement de l'intérêt communautaire redonnerait aux communes la liberté de décider des zones d'activités pour lesquelles l'échelon communautaire serait le plus pertinent et de celles qui pourraient rester dans le giron communal. La

le transfert aux communautés urbaines et aux métropoles des compétences création, aménagement et entretien de la voirie, signalisation, abris de voyageurs et parcs et aires de stationnement, d'autoriser la restitution aux communes membres de ceux qui ne seraient pas jugés tels ». Cela signifie que les

pour présenter l'amendement n° 565 rectifié. La commission des lois a modifié les modalités de la définition de l'intérêt communautaire pour l'ensemble des strates d'intercommunalité- communautés de communes, communautés d'agglomération, communautés urbaines et métropoles. Désormais, le vote requis pour définir l'intérêt communautaire ou métropolitain s'effectuerait à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, et non plus à la majorité des deux tiers des membres du conseil. Au vu des compétences exercées par les communautés urbaines et les métropoles, plus haut niveau d'intégration intercommunale en France, cette définition constitue un enjeu majeur. Elle doit donc faire l'objet d'une véritable majorité, qui ne saurait se limiter aux seuls suffrages exprimés. Cet amendement vise donc à en rester au droit en vigueur pour les communautés urbaines et les métropoles : l'intérêt communautaire et métropolitain est déterminé à la majorité des deux tiers des membres du conseil, et non des suffrages exprimés. La parole

de l'intérêt communautaire ou métropolitain et délimiter ainsi les compétences transférées au niveau intercommunal est la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, et non pas

dans la proposition de loi visant à encourager l'adoption de règlements locaux de publicité intercommunaux. Sans garantie sur l'inscription de cette proposition de loi à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, mon amendement vise à les introduire dans le présent projet de loi.

puisque les anciens RLP, adoptés avant 2010 par plus de 1 200 communes, seront frappés de caducité au 14 juillet 2020. De plus, les ajustements relatifs à l'élaboration et la modification des PLU apportés par la loi de 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté

La proposition de loi que j'ai déposée en avril 2019, complétée lors de son examen par la commission des affaires économiques, et adoptée par le Sénat le 1 octobre dernier, comporte quatre mesures. Elle valide les RLP intercommunaux élaborés selon les procédures assouplies applicables au PLU. Elle confirme que ces procédures leur sont bien applicables

Avec le report de la caducité, il est nécessaire de décaler également cette entrée en vigueur. Enfin, elle instaure pour les tiers un délai de mise en conformité avec les nouvelles réglementations qui s'appliqueront après la caducité des RLP de première génération.

un véhicule législatif dans le délai nous permettant de le voter avant la date de caducité, à savoir le 14 juillet 2020. Nous sommes très heureux que cet amendement puisse être intégré

restons dans le même domaine, puisque cet amendement vise à sécuriser la situation juridique des EPCI à fiscalité propre auxquels les communes ont transféré la compétence pour édicter un règlement local de publicité, sans leur transférer la compétence en matière de PLU.

Aussi rassurante soit-elle, une telle réponse n'a pas une portée suffisante pour empêcher l'annulation d'un RPL intercommunal en cas de contentieux. Le présent amendement vise donc à clarifier les choses. Il tend à s'inscrire dans la droite ligne de la volonté du Sénat d'écrire un droit plus lisible.

d'un amendement porté par Jean-Yves Roux. Les élus, en particulier ceux des petites communes, sont interpellés régulièrement, mais surtout directement, par nos concitoyens. C'est non pas la présidente ou le président de l'intercommunalité, mais le ou la maire de sa commune qui doit répondre à tant d'interpellations sur ce qui se passe dans le périmètre de la commune. Or les modalités de transfert de compétence échappent à la plupart des administrés. Dans les faits, les transferts obligatoires de compétences, et en particulier les compétences morcelées - je pense à la compétence scolaire -, n'enlèvent rien aux missions essentielles des communes au service de la cohésion sociale et de la qualité de vie de nos concitoyens. Il s'agit donc de traduire dans la loi les pratiques démocratiques vécues par nos concitoyens. Enfin, dans un contexte où tant de maires hésitent à s'engager de nouveau, il nous paraît indispensable de rappeler que la commune, bras armé de la proximité, constitue bien, selon la formule consacrée, la cellule de base de la démocratie locale.

une disposition figurant dans la proposition de loi de nos collègues Bas, Retailleau et Darnaud, qui portait sur l'équilibre territorial et la vitalité de la démocratie locale. Depuis sa mise en oeuvre en 2017, la carte des EPCI à fiscalité propre propre a atteint ses objectifs, à savoir la couverture totale du territoire national et l'agrandissement des intercommunalités. Elle est censée présenter une certaine stabilité. Les modifications de la carte doivent désormais s'opérer sur la base d'une démarche volontaire des élus, en lien avec les préfets,

aux seuils de population, à la cohérence sociale, spatiale, ou encore à la solidarité financière et territoriale, doivent néanmoins être conservées au titre des objectifs de l'organisation de la carte intercommunale. intercommunale, la CDCI, le cas échéant, puisse en tenir compte dans ses observations, puisqu'elle tient à jour un état de la coopération intercommunale dans les départements. Il s'agit donc d'une mesure de simplification.

le document existant sert encore de référence pour un certain nombre de sujets, notamment la création éventuelle de syndicats de communes ou de syndicats mixtes, avec la procédure de fusion-extension qui pourrait s'appliquer. Par ailleurs, le schéma détermine le champ de l'obligation de consultation de la CDCI. Je propose que le droit reste en l'état.

naturellement difficile à réunir en raison d'une emprise préfectorale parfois très forte sur les communes. La commission se prononce ensuite sur le schéma par un avis qui ne lie pas le préfet. Ainsi, actuellement, un préfet peut valider un schéma départemental sans que celui-ci ait été approuvé par la CDCI. Le présent amendement vise à redonner un pouvoir accru à la commission, en imposant au préfet de soumettre le projet de schéma à son approbation à la majorité des deux tiers.

qui ont imposé des unions forcées. Toutefois, mon cher collègue, votre amendement ne tend pas à supprimer la disposition selon laquelle la CDCI est réputée favorable si elle ne s'est pas prononcée dans un délai de trois mois.

Dans d'autres cas, on a assisté à des fusions opérées par des élus qui avaient un peu de poids politique et qui ont procédé à des extensions brutales. Dans mon département, certaines grandes intercommunalités

que le service public se soit développé avant même l'apparition de l'intercommunalité dans notre pays ! Dès l'après-guerre, on a su amener l'électricité jusqu'à la ferme la plus isolée grâce à un système de péréquation. La question

départementaux de coopération intercommunale, conformément à la loi NOTRe, a entraîné un profond bouleversement du fonctionnement des EPCI, dont les périmètres et les compétences ont été élargis. Cette réorganisation, réalisée parfois dans des conditions difficiles, a pu aboutir à des structures dont l'efficacité pose question et dont le fonctionnement s'avère insatisfaisant pour les élus municipaux. S'il est nécessaire d'apporter des réajustements aux périmètres des EPCI, il faut éviter que ceux-ci ne se produisent au fil de l'eau, avec des changements réguliers de périmètre, qui ont pour conséquences de déstabiliser les EPCI et d'amoindrir la visibilité, notamment financière, nécessaire à leur gestion. C'est pourquoi le présent amendement, proposé par le président Hervé Maurey, tend un nouveau dispositif prévoyant une échéance à mi-chemin de la prochaine mandature, au 30 juin 2023, pour réaliser un bilan de fonctionnement et, si besoin, faire évoluer les périmètres des EPCI. Jusqu'à cette date, il ne pourra plus être procédé à des changements de périmètre d'EPCI, si ce n'est à des créations d'EPCI par partage d'EPCI existant, telles qu'elles sont prévues à l'article 10 du présent texte, que nous n'avons pas encore examiné. Ce bilan peut contenir des préconisations relatives au périmètre de l'EPCI. Après accord des conseils municipaux concernés par le retrait, les propositions de retrait sont effectuées dans le cadre des procédures simplifiées de retrait applicables aux communes quittant une communauté de communes et, aux termes du présent texte, aux communes quittant une communauté d'agglomération. Cet amendement a pour objet que l'adhésion des communes au nouvel EPCI s'effectue dans le cadre du droit commun. Dans le cas où le retrait aurait pour but un partage de l'EPCI en plusieurs EPCI, la procédure applicable est celle qui est prévue à l'article 10 du présent texte, que nous n'avons pas encore examiné.

obliger chaque intercommunalité à réaliser, au plus tard le 30 juin 2023, un bilan qui conditionnera des évolutions de périmètre me semble contrevenir à l'urgence de procéder à des modifications de périmètre qui devraient pouvoir être actées assez rapidement. Je vous rappelle que, dans ce texte de loi, nous proposons

un certain nombre d'élus de notre sensibilité politique ont toujours défendu, sur l'ensemble du territoire national, la création

Cette décision doit être actée par l'ensemble de parties prenantes. Comme il y a des mariages réussis, il y a des divorces réussis !

que la procédure de droit commun. Or vous nous proposez d'appliquer à la procédure de retrait dérogatoire des conditions plus difficiles que les règles de droit commun.

Le présent amendement vise à supprimer le seuil de création démographique- 250 000 habitants -pour les communautés d'agglomération qui souhaiteraient se transformer en communauté urbaine. En effet, le poids démographique ne dit rien du niveau d'intégration d'une intercommunalité, de la maturité d'une histoire commune, ni du souhait de son exécutif, démocratiquement élu, de remplir les responsabilités d'une communauté urbaine, telles qu'elles sont définies par la loi : un « espace de solidarité, pour élaborer et conduire ensemble un projet commun de développement urbain et d'aménagement de leur territoire. il est proposé de permettre à des territoires ne remplissant pas les conditions de population actuelles- 250 000 habitants - de poursuivre leur dynamique commune d'intégration de compétences et de construction d'un projet de territoire, qui ne se limite d'ailleurs pas à leurs seules frontières administratives. En effet, les communautés urbaines, par les compétences qu'elles exercent, assument aujourd'hui un rôle structurant à l'égard des territoires voisins, dans une logique de coopération et d'alliance des territoires. Il importe donc de ne pas freiner les logiques d'intégration et de coopération en figeant des critères purement démographiques qui nuiraient à la mise en capacité des territoires, laquelle se révèle évolutive. En proposant de supprimer le seuil démographique, le présent amendement peut potentiellement permettre, en l'état actuel de la carte intercommunale, à 27 communautés d'agglomération supplémentaires d'accéder à un statut constitutif d'une libre volonté de plus grande maturité intercommunale. On rappellera enfin que depuis la réforme de la dotation d'intercommunalité- c'est l'article 250 de la loi de finances pour 2019

tend à redonner aux communes une forme de liberté et à élargir aux communes membres d'une communauté urbaine la procédure de retrait de droit commun. Cette procédure, prévue à l'article L. le CGCT, autorise le départ d'une commune, sous réserve de l'accord de l'organe délibérant de la communauté de communes. Cette extension aux communes membres de communautés urbaines permettra la mise en oeuvre, localement, d'ajustements des schémas départementaux de coopération intercommunale.

Merci,